de la commission

Mme le rapporteur. Cet amendement vise à abroger une disposition prévoyant la remise d'un rapport par les organisations liées par une convention de branche sur les écarts de rémunération entre femmes et hommes. Ce rapport n'a pas lieu d'être en raison de la nouvelle obligation qui leur est imposée d'établir un bilan annuel de leurs actions en faveur de l'égalité professionnelle.

n° 647 Il s'agit d'un amendement de coordination juridique. Depuis la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, les entreprises qui n'auraient pas satisfait à leur obligation de négocier en matière d'égalité professionnelle doivent être exclues de la procédure de passation des marchés publics. Cette interdiction de soumissionner a été reprise dans l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et dans l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Cependant, ces ordonnances font encore référence à l'ancien article L. 2242-5 du code du travail. la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, puis l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ont modifié les dispositions relatives à l'obligation de négocier en matière d'égalité professionnelle. Il est donc nécessaire de mettre à jour les références à l'article du code du travail concerné dans ces deux ordonnances afin de redonner une base légale à cette disposition.

Le projet de loi prévoit un certain nombre de mesures visant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes. La plupart

d'être sensibilisé à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle leur permettra également de prendre conscience de l'impact que des projets apparemment neutres peuvent avoir. On le sait, des dispositions, des critères ou des pratiques apparemment neutres peuvent entraîner un désavantage particulier pour certains groupes de personnes. C'est ce qui s'appelle la discrimination indirecte. L'intervention des institutions représentatives du personnel sur chaque grand projet permettra de lutter en amont sur les discriminations indirectes, qu'elles soient volontaires ou non. Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons l'introduction d'un nouvel alinéa à l'article L. 2312-8 du code du travail.

ne pourrait être plus de vingt fois inférieur à la rémunération annuelle globale la plus élevée, que celle-ci soit celle versée à un salarié ou à un dirigeant mandataire social non salarié. Cet encadrement aurait ainsi vocation à remplacer le plafond de rémunération de 450 000 euros mis en place dans les entreprises publiques. Nous répétons

l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette sanction consisterait en la suppression d'une exonération de cotisations sociales patronales pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations. Depuis les années 2000, une vingtaine de lois traitant de l'égalité entre les femmes et les hommes ont été adoptées, dont une dizaine portaient spécifiquement sur l'égalité au travail.

à 19 %. Si les inégalités persistent, c'est parce qu'il n'existe pas de sanction systématique et suffisamment sévère incitant les entreprises à respecter leurs obligations. C'est pourquoi nous proposons d'assortir d'une sanction les obligations des entreprises en matière de négociation sur l'égalité professionnelle. Actuellement, le code du travail impose une négociation sur l'égalité tous les quatre Lorsque cette négociation n'aboutit pas à la conclusion d'un accord collectif, l'employeur a l'obligation d'établir unilatéralement un plan d'action annuel, destiné à assurer l'égalité professionnelle. Pourtant, 60 % des entreprises assujetties à cette obligation n'ont ni conclu un accord ni établi un plan d'action. Et seules 0,2 % d'entre elles ont été sanctionnées ! Afin de faire respecter cette obligation, nous proposons que les entreprises ne disposant

j'invite le Gouvernement à préserver les compétences déjà existantes en matière d'accompagnement des femmes victimes de harcèlement ou de discriminations professionnelles. Je pense particulièrement à l'AVFT,

confortée dans sa capacité à répondre aux besoins des femmes victimes de harcèlement ou de discriminations salariales. Par ailleurs, j'ai vu l'appel d'offres qui a été lancé, je vois le choix qu'est en train de faire le Gouvernement. Je rappelle donc que, sur ces sujets, on ne s'improvise pas du jour au lendemain référent, accompagnant ou expert juridique auprès des femmes et que les compétences qui existent, qui ont été construites après des années de travail, comme celles de l'AVFT, doivent être préservées et encouragées.

Le harcèlement et les agressions sexuelles au travail touchent plus d'un tiers des femmes au travail. Certes, la création des référents chargés, dans les entreprises, d'orienter et d'accompagner les victimes ne permettra pas de résoudre tous les problèmes.

servir de relais indépendants à même d'écouter et d'aider les victimes. Il ne s'agit aucunement de revenir sur les obligations des employeurs en matière de sécurité physique et psychique des salariés ou sur les pouvoirs disciplinaires des employeurs. Il faut par ailleurs savoir raison garder, les référents ne fonctionneront pas pas en autarcie complète. Ils travailleront de concert avec les employeurs. L'enjeu est ici de définir un relais connu de tous. Je le dis avec gravité, il ne faut ni surestimer ni sous-estimer cette mesure. Non,

espace de vie central au quotidien. J'ajoute que la destruction à petit feu de l'inspection et de la médecine du travail, réforme après réforme, réduit encore les possibilités d'action de ces structures pour lutter efficacement contre les risques

vient de défendre Mme Assassi. La lutte contre le harcèlement sexuel ou sexiste dans l'entreprise, comme celle pour l'égalité salariale, est beaucoup moins consensuelle dans la réalité l'on pourrait l'imaginer ou le croire. Les stratégies de résistance sont encore développées dans un certain nombre d'entreprises. Il suffit d'ailleurs de consulter le bilan des entreprises du SBF 120 pour voir qu'il existe de grandes disparités dans la manière dont elles

les prérogatives du référent en charge de la lutte contre le harcèlement : droit d'assister une éventuelle victime, droit d'alerte, droit d'être informé des étapes et du contenu de la procédure d'enquête, droit d'accompagner l'inspection du travail, droit de saisine de l'inspection du travail, droit de saisine et inscription d'une question à l'ordre du jour du comité social et économique de l'entreprise.

susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes, le refus de l'employeur devant être motivé. En la matière,

la peur au ventre quand elles vont au travail, comment voulez-vous qu'elles se projettent dans l'avenir professionnel ? On ne peut pas, d'un côté, vouloir l'égalité professionnelle des salaires et des carrières, et, de l'autre, ne pas prendre en compte un tel phénomène. Force est

En ce qui concerne l'amendement n° 592, j'y suis également favorable sur le principe, pour les raisons que je viens d'expliquer. En revanche, il n'est pas nécessaire de préciser les prérogatives dont le référent dispose en matière d'alerte, de saisine de l'inspection ou encore d'assistance aux victimes, puisque celles-ci sont déjà celles d'un délégué du CSE.

Cet amendement vise à prévoir que tout signalement de harcèlement sexuel au travail transmis aux agents de l'inspection du travail doit faire l'objet d'une enquête par ces mêmes agents. Nous avons trop d'exemples,

admet, depuis plusieurs années, que le licenciement d'une salariée pour dénonciation de faits de harcèlement sexuel est nul de plein droit, sauf à ce que l'employeur puisse démontrer la fausseté de ces allégations, et ce quand bien même d'autres motifs de licenciement auraient été mentionnés dans la lettre de licenciement. Ces motifs complémentaires n'ont pas à être examinés, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que le licenciement a été d'une victime de faits de harcèlement. La législation récente, par le biais des ordonnances, est revenue sur cette jurisprudence, juste et constante, de la chambre sociale de la Cour de cassation, alors même que les licenciements intervenus pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sont assez rares, les employeurs utilisant, en général, d'autres motifs pour licencier ces salariés. Aussi, l'intérêt patronal de ces dispositions est, quoi qu'il en soit, minime. Cet amendement vise donc à revenir sur ce qui avait été décidé au travers des ordonnances et à rétablir,

ayant souhaité alerter la direction de l'entreprise sur des actes dont il a été témoin sera annulé par le conseil de prud'hommes. Le premier alinéa de l'amendement, outre qu'il tend à introduire l'innovation d'une présomption subséquente à un jugement, se trouve donc satisfait par le droit en vigueur. Le second, en tant qu'il porte une atteinte manifeste à la séparation des pouvoirs,

également été formulée par le Défenseur des droits. Dans la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a été votée une disposition prévoyant que l'indemnisation du préjudice liée à la rupture du contrat de travail

prévu par les ordonnances est défavorable aux victimes de harcèlement ou de discrimination. ? Avis défavorable. Ce débat a déjà eu lieu dans l'hémicycle, lors de la ratification des dernières ordonnances Travail. Notre assemblée s'était alors prononcée pour une harmonisation du plancher à six mois pour toutes les indemnisations pour licenciement abusif.

Cet amendement vise à renforcer la prise en charge de la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles dans le cadre de la négociation collective. Il est inspiré par des préconisations portées par des spécialistes de l'égalité professionnelle,

Inclure cette dimension permettrait en outre de donner une concrétisation supplémentaire à la grande cause nationale voulue par le Président de la République.

Cet amendement vise à diminuer la périodicité à laquelle sont négociés les thèmes relatifs aux salaires, aux mesures tendant à favoriser l'égalité professionnelle, aux conditions de travail, à la situation des personnes handicapées et au régime de formation professionnelle.

La parole est à Mme Laurence Rossignol. Cet amendement vise à sanctuariser, au sein de la négociation collective, la préservation des droits familiaux et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

la France accuse un retard par rapport à ses voisins. Une réforme du congé de paternité constituerait un levier essentiel pour réduire les inégalités professionnelles. Aujourd'hui, les pères bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze jours consécutifs, qui s'ajoute au congé de naissance de trois jours. Ce congé est optionnel. Rappelons que le taux de recours au congé de paternité n'est que de 68 %. Pourtant, les comparaisons européennes montrent que, dans les pays où la législation promeut des congés parentaux plus longs et parfois obligatoires, les inégalités se réduisent et une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle est constatée. C'est notamment observable au Portugal, où les pères ont droit à un mois de congé de paternité, dont deux semaines obligatoires. Le Gouvernement a récemment rejeté l'idée de rendre obligatoire le congé de paternité. Pourtant, sur les seize semaines de congé de maternité, huit sont obligatoires, dont six après la naissance, afin de s'assurer que l'employeur ne fait pas pression sur sa salariée pour qu'elle ne prenne pas le congé auquel elle a droit. Pourquoi en serait-il autrement pour les hommes ? Le taux de non-recours de 32 % au congé de paternité s'explique notamment par la pression professionnelle subie. Il est donc indispensable de garantir ce droit en le rendant obligatoire. Cet amendement est une première étape

Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à rééquilibrer entre les deux parents l'impact d'une naissance sur la carrière et à réduire les inégalités professionnelles, en donnant la possibilité au père de s'impliquer un peu plus dans les premiers jours qui suivent la naissance de l'enfant. En matière d'égalité professionnelle et de partage des tâches, nous sommes loin du compte. Il est donc indispensable de revoir la durée des congés, notamment du congé de paternité. Aujourd'hui, les pères bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze jours consécutifs, qui s'ajoute au congé de naissance de trois jours accordé et rémunéré par l'employeur. l'article 40 de notre Constitution ne nous permet pas d'allonger le congé de paternité. Seul le congé de naissance peut l'être, car son financement est à la charge du seul employeur. C'est pourquoi nous proposons, par cet amendement, d'allonger le congé de naissance de trois Pourquoi dix-sept ? Parce que cela permettrait de doubler la durée cumulée actuelle du congé de naissance, trois jours, et du congé de paternité, onze jours, en la passant de quatorze Rappelons que, pour rejeter le droit individuel à un congé parental d'au moins quatre mois, contenu dans le projet de directive sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants, actuellement en discussion au Parlement européen, le Gouvernement a avancé des arguments de coût budgétaire et a indiqué qu'il préférerait allonger le congé de paternité. J'espère que le Gouvernement fera preuve de cohérence et émettra un avis favorable sur cet amendement.

à plusieurs titres. Premièrement, on ne peut que s'interroger sur la pertinence de l'introduction dans ce texte de tels dispositifs de pantouflage. Il y a fort à parier que, si ces mesures avaient été proposées par un groupe parlementaire, elles auraient été rejetées en tant que cavaliers législatifs. Ces suppressions sont donc signe de cohérence. Deuxièmement, et c'est le plus important, cette volonté gouvernementale de promouvoir le pantouflage témoigne de deux volontés convergentes. La première

de caste, un groupe réduit d'individus naviguant dans ce que j'appelle le « pouvoir caché ». Car, soyons sérieux, lorsque l'on parle de pantouflage, on ne parle pas d'un aide-soignant devenu restaurateur. Comme l'a montré notre collègue Pierre-Yves Collombat, si le pantouflage est minoritaire dans la fonction publique, il se concentre dans certains secteurs.

L'argument avancé par le Gouvernement de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas satisfaisant. S'il est vrai que les femmes demandent plus souvent une mise en disponibilité que les hommes, ce sont ces derniers qui sollicitent le plus des mises en disponibilité de convenance, dans le champ d'application des articles concernés. Clairement, ce cynisme et cette instrumentalisation n'honorent pas le Gouvernement. La suppression des articles était un premier pas, mais le problème du pantouflage demeure. nous vous proposons de franchir le gué en interdisant à un agent public devenu lobbyiste de mener son activité auprès de ses anciens collègues, et ce dans un souci de lutte contre les conflits d'intérêts et la collusion que peuvent engendrer des années de travail en commun.

durant laquelle un fonctionnaire ayant quitté la fonction publique ne peut pas mener des opérations de lobbying auprès de son administration de rattachement. On le sait, les agents publics, et surtout les hauts fonctionnaires, font l'objet d'une cour assidue, quand ce ne sont pas les institutions mêmes qui les poussent dans les bras du privé. Ainsi, la mission de suivi personnalisé des parcours professionnels, à Bercy, va jusqu'à recenser les offres d'emploi du privé pour les mettre à disposition des cadres du ministère. En parallèle, la capacité d'action de la commission de déontologie et de contrôle demeure assez floue. Pour ne prendre qu'un exemple, cette commission a quand même réussi à valider la nomination, le 2 mars 2009, d'un fonctionnaire à la tête de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de la Banque fédérale des banques populaires, moins d'une d'une semaine après que celui-ci eut organisé la fusion de ces deux organismes. Ces pratiques d'un autre temps remettent totalement en cause le principe même de la fonction publique, fondée sur le mérite républicain. Je me permets une légère digression pour rappeler que le recrutement au concours des fonctionnaires a été une mesure de progrès social visant à replacer le mérite au premier plan, au détriment du népotisme qui existait jusque-là.

Ce constat d'une reproduction sociale tient à deux éléments : l'incapacité de l'école républicaine à gommer les inégalités de capitaux et le recrutement d'entrée à l'ENA, qui se fait à plus de 80

Le mécanisme que nous proposons, s'il ne permet pas de lutter totalement contre ce phénomène, vise à créer une période tampon de dix ans durant laquelle un ancien fonctionnaire ne peut faire du lobbying auprès de son administration de rattachement, c'est-à-dire concrètement auprès de ses anciens collègues. L'enjeu est bien de préserver autant que possible

à des demandes de disponibilité pour convenance personnelle, notamment liées à la naissance d'un enfant après un congé parental- que l'on s'en réjouisse ou pas, la société est ainsi faite aujourd'hui que les demandes sont plus souvent portées par des femmes que par des hommes dans ce cas-là -ou à des

très souvent une femme, demande un congé parental, son avancement de carrière est protégé la première année, mais réduit de 50 % la deuxième et troisième année. Dans le cadre du renouvellement de l'accord sur l'égalité salariale femmes-hommes dans la fonction publique- nous espérons qu'il pourra être renouvelé à la rentrée, autour du mois d'octobre -, nous avons élargi nous avons élargi les champs de l'accord à la question de la maternité et de la parentalité pour faire en sorte, comme nous le proposons dans le cas des disponibilités pour expérience professionnelle dans le privé, de garantir l'avancement de carrière au moins pendant le congé parental, et peut-être aussi pendant les deux premières années

Cette commission d'enquête doit prendre fin en septembre et devrait émettre des recommandations. Je trouve bizarre

qui brouille, une fois de plus, les lignes entre le public et le privé et qui favorise de nouveau l'immixtion des intérêts privés dans la sphère publique. Sans préjuger des conclusions de la commission d'enquête du Sénat sur les mutations de la haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de

comme cela a été dit, ils n'ont fait l'objet d'aucune concertation, ni avec les représentants des employeurs publics ni avec les organisations syndicales ou associations professionnelles, alors même que des négociations viennent d'être ouvertes en vue d'un projet de loi relatif à la fonction publique en 2019. Ces amendements

de disponibilité pour exercice dans le privé ont été examinées par le Conseil commun de la fonction publique, au moins de mars, avec un avis favorable du collège des employeurs et un avis plus partagé du collège des organisations syndicales, certaines organisations parfois qualifiées de réformistes s'étant toutefois prononcées en faveur de ces dispositions.

question de dévoiler les travaux d'une commission d'enquête. Je suis bien placée, comme présidente de groupe, pour affirmer que je respecte les travaux de toutes

fait courir pour la gestion des administrations publiques des risques sans précédent. Force est de constater que le recrutement par contrat de hauts fonctionnaires, aujourd'hui possible, mais dérogatoire, deviendrait inexorablement le mode de recrutement

proclamé par l'article VI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le principe de l'égale admissibilité aux emplois publics est unanimement reconnu comme la pierre angulaire du droit de la fonction publique. De plus, cette évolution, faussement présentée dans les médias comme concernant uniquement la haute fonction publique, a en réalité un impact sur l'ensemble de la fonction publique et de son encadrement supérieur.

cet amendement, qui a pour objet de pallier les difficultés rencontrées en matière de recrutement dans des établissements publics dont le personnel relève de la fonction publique hospitalière. Cette disposition permet un recrutement de contractuels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, en l'absence de candidat fonctionnaire titulaire.

à vous remercier

Cela est d'autant plus paradoxal que les concours internes sont ouverts aux personnes qui ont accompli des services au sein des administrations, organismes et établissements des autres États membres membres de l'Union européenne ou États parties à l'Espace économique européen. Autrement dit, si vous êtes Français, vous ne pouvez pas vous présenter, mais si vous êtes italien et avez travaillé dans une ambassade italienne, vous pouvez vous présenter. C'est tout de même une situation étonnante ! Il semble que le Gouvernement envisage d'autoriser les recrutés locaux à se présenter aux concours Une telle décision irait dans le bon sens, mais le nombre de places offertes selon cette procédure est très inférieur à ce qui se pratique pour les concours internes. De plus, la troisième voie est ouverte à des personnes disposant d'une expérience professionnelle dont la durée est plus longue que celle qui est exigée pour se présenter à un concours interne. Pour toutes ces raisons, nous proposons d'ouvrir les concours internes aux recrutés locaux, en sus de l'ouverture des troisièmes concours. Nous souhaitons ainsi permettre aux corps de fonctionnaires du ministère de l'Europe et des affaires étrangères de bénéficier des compétences des agents de droit local

Les agents de droit local ne sont pas des agents de droit public et ouvrir un concours interne à ces agents viendrait bousculer l'équilibre des concours internes. Nous avons travaillé à une solution alternative, que vous avez évoquée : ouvrir se présenter aux concours dits de la troisième voie à l'ensemble des agents recrutés en droit local, qu'ils soient de catégorie A, B ou C. Je puis vous affirmer que, d'ici à la fin de l'année 2018, l'intégralité des métiers et des corps seront couverts par cette possibilité d'accès à la titularisation par la troisième voie. En cela, votre amendement me semble satisfait. Il l'est d'autant plus que nous avons veillé,

Au-delà des motifs indiqués dans l'objet de cet amendement, il est notable que ces mesures, si elles étaient votées, entraîneraient une transformation majeure de l'organisation des collectivités, sans que l'impact en soit mesuré à ce jour.

Considérer que tous les postes dirigeants peuvent être occupés par un contractuel, y compris dans les collectivités de petite dimension, c'est considérer que le rôle des directeurs généraux est dénué de lien avec les responsabilités régaliennes que les collectivités mettent en oeuvre au quotidien aussi considérer que la gestion des collectivités ne fait pas appel, jour après jour, aux prérogatives de puissance publique au travers de ses fonctionnaires. Ce serait le premier pas vers une sorte de désacralisation du rôle même des collectivités dans le modèle français.

des fonctionnaires et de conforter leurs spécificités et leur capacité à gérer la complexité, fruits d'un apprentissage que l'université ne permet pas. Leur expertise est appréciée, recherchée par les associations d'élus. La présence généralisée de dirigeants contractuels exposera la collectivité à des conflits d'intérêts potentiels plus nombreux et à des conséquences pénales importantes. Elle soumettra ces postes à une pression politique accrue, là où le statut a jusqu'à présent joué un rôle de garde-fou. Il n'est nul besoin de recrutements politisés pour bien mettre en oeuvre les projets politiques ; loyauté et neutralité ne peuvent s'opposer. Ces principes sont le ciment du lien de confiance entre les élus et les cadres dirigeants. Ce lien qui existe entre un exécutif et sa direction générale est complexe et ténu, il fonde une grande partie de la légitimité du dirigeant. Il est bon de rappeler qu'avant 1946- dans l'ancien monde ... -il n'y avait que peu de règles et pas de réel statut. Chacun pouvait être recruté dans un service public. Les historiens peuvent nous éclairer, sans remonter aux fermiers généraux, sur les dérives de la privatisation de la chose publique, à l'échelon tant national que local. Avant la mise en place du statut, le clientélisme politique existait largement.

de formation des apprentis, CFA, aux branches professionnelles est dangereux pour l'avenir de nos jeunes dans la mesure où, faute d'être suffisamment structurées, ces dernières sont incapables d'assumer seules cette compétence.

La valorisation du compte personnel du salarié en euros n'est pas adaptée aux coûts unitaires moyens complets des formations financées. Le différentiel de coût horaire est de l'ordre de 30 % par rapport aux coûts pratiqués dans l'Hexagone. Enfin, dans certains territoires, le financement de la formation fait peser des risques sur le statut juridique et la pérennité de certains établissements : je pense à Guadeloupe Formation, créé par le conseil régional et récemment transformé Ce constat, partagé par le président de l'Association des régions de France et par le Gouvernement qui a proposé, lors de l'audition de Mme la ministre par la commission, puis par la délégation aux outre-mer à l'Assemblée nationale, d'identifier les adaptations nécessaires, nous a amenés à proposer des amendements collant à la réalité et aux besoins de nos territoires ultramarins. À cette heure, nous attendons toujours le projet d'ordonnance promis par Mme la ministre lors de nos différents échanges et destiné à procéder aux adaptations nécessaires. Si nous contestons la méthode qui consiste, une fois de plus, à donner un blanc-seing au Gouvernement pour légiférer à notre place, nous souhaitons que le plus grand nombre d'acteurs soient consultés et associés à l'élaboration de la future ordonnance et des décrets d'application. C'est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement, que l'élaboration de l'ordonnance prévue par le présent article prenne en compte les caractéristiques et contraintes particulières des collectivités concernées, termes reconnus constitutionnellement et sur lesquels se fondent l'ensemble des adaptations législatives pour les outre-mer. Il s'agira de faire en sorte que l'ordonnance prenne concrètement en compte le bas niveau de formation initiale sur ces territoires,

Le CDI intérimaire, introduit à titre expérimental et intégré à la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, connaît, depuis sa mise en place, un fort développement.

gagnant pour le salarié, qui bénéficie d'un cadre contractuel fixe qui réduit sa situation de précarité et permet d'assurer son employabilité grâce aux formations qui lui sont dispensées gagnant pour l'entreprise de travail temporaire, puisque le dispositif lui permet de continuer à offrir à ses clients la flexibilité attendue, tout en répondant à leurs besoins actuels et futurs en termes de compétences. Depuis sa mise en place, ce dispositif a incontestablement permis une intégration durable dans l'emploi de travailleurs temporaires et s'est révélé un outil efficace contre la précarisation des salariés. Il gagnerait donc à être pérennisé, ce qui passe par son inscription dans le code du travail. Quel est l'avis

du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Son adoption complétera notre approche d'une flexisécurité à la française, qui vise à sécuriser les parcours et à lutter contre la précarité excessive, tout en permettant aux entreprises d'être agiles.

nationale et au Sénat, de nombreux amendements ont été examinés visant à demander des rapports sur les différents volets de ce projet de loi, marquant ainsi la volonté des parlementaires d'en suivre l'application.

un comité de suivi chargé de l'application de la présente loi, qui garantira aux parlementaires un droit de regard et d'évaluation continu. Très bien

la gestion de la formation professionnelle a été régionalisée, afin d'adapter le plus possible la formation aux exigences des entreprises, dans un but d'employabilité et au détriment de l'acquisition de diplômes et de qualifications. En matière d'assurance chômage, le Gouvernement a instauré sa mainmise sans tenir ses promesses. En effet, le passage d'un financement par les cotisations à un financement par l'impôt ainsi que le cadrage de la négociation de la convention UNEDIC permettent au Gouvernement de prendre le contrôle de l'assurance chômage. l'ouverture de l'allocation chômage aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants est encadrée dans des conditions tellement strictes que l'on estime qu'elle ne bénéficiera qu'à 50 000 personnes au maximum, bien loin de la promesse d'universalité du Gouvernement. Enfin, le volet du projet de loi portant des dispositions diverses relatives à l'emploi s'est révélé décevant. Certes, de nombreuses mesures relatives aux travailleurs handicapés et en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ont été adoptées, mais aucune des propositions visant à mieux protéger les travailleurs des plateformes n'a été retenue. Pendant les débats, notre groupe a défendu un projet alternatif, comme nous avons l'habitude de le faire pour chaque texte examiné. Celui-ci reposait, d'une part, sur un service public national de l'enseignement, ayant pour objectif l'acquisition de qualifications et non l'employabilité, et, d'autre part, sur la sécurisation des parcours professionnels des actifs, grâce à l'instauration d'une allocation autonomie jeunesse et à la création d'une sécurité sociale réellement universelle. Ce texte étant l'exact opposé du projet que nous avons défendu, nous voterons contre.

sociales favorables aux salariés ou aux demandeurs d'emploi. Ce n'est plus le cas en 2018 : le big bang conduit le Gouvernement à proposer un texte en opposition avec plusieurs choix affirmés par les partenaires sociaux. Stupéfaction,

c'est bien la première fois qu'une compétence confiée aux régions depuis 1981-1983 est remise en cause au bénéfice des branches professionnelles et de l'initiative privée, au risque de creuser les inégalités entre les territoires et les secteurs d'activité. seconde rupture a trait à la nouvelle gouvernance par une institution publique quadripartite : France compétences, qui n'a fait l'objet d'aucune négociation et qui affaiblit considérablement l'un des trois piliers du du paritarisme. Il semble bien que le Président de la République n'aime pas les corps intermédiaires, ce qui n'est pas un bon signe au moment d'engager la réflexion sur une nouvelle sécurité sociale. D'autres points de désaccord

prendre des décisions aussi importantes pour l'avenir de notre pays

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.